La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 25 juin 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? Le procès-verbal est adopté. M. Christophe Chaudun a fait connaître à M. le président du Sénat qu'il se démettait de son mandat de sénateur de la Sarthe à compter du jeudi 25 juin 2020, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par Mme Muriel Cabaret, dont le mandat de sénatrice a commencé vendredi 26 juin, à zéro heure. En application des articles L.O. 151 et L.O. 297 du code électoral, M. le président du Sénat a pris acte de la fin de plein droit, à compter du samedi 27 juin, à minuit, du mandat de sénateur de l'Ardèche de M. Jacques Genest. En application de l'article L.O. 319 du code électoral, il est remplacé par Mme Catherine André, dont le mandat de sénatrice a commencé dimanche 28 juin, à à zéro heure. En votre nom à toutes et tous, je souhaite la plus cordiale bienvenue à nos nouveaux collègues. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires sociales a été publiée. Elle sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. règlement. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale

et, je l'espère, adopter cette proposition de loi revalorisant les pensions de retraite agricoles, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale sur la proposition du député André Chassaigne. ; tout d'abord, parce qu'il s'agit d'une question de justice sociale ; ensuite, parce que le travail et la production des agriculteurs sont essentiels pour notre pays et pour chacun d'entre nous parce que le niveau des pensions agricoles n'est pas digne du travail de ces acteurs indispensables pour nos territoires. Mesdames, messieurs les sénateurs, le système de pensions agricoles est issu d'une longue et riche histoire. illustre l'évolution des activités dans notre pays. Il pose la question de notre engagement, en tant que société, vis-à-vis de cette profession universelle. Nos agriculteurs ne nous demandent pas l'aumône : ils ont droit à la reconnaissance de chacun d'entre nous. Et ils ont surtout le droit d'avoir la garantie d'une vie digne quand l'âge ne rend plus possible la poursuite de l'activité professionnelle. Mesdames, messieurs les sénateurs, la situation des retraités agricoles nous parle aussi d'universalité et de solidarité. Je voudrais souligner qu'il y a là comme un paradoxe : le système de retraite agricole est catégoriel.

Ces régimes à points fonctionnent grâce à la solidarité nationale, car les deux sont bien compatibles, pour ceux qui en douteraient ... Je sais, mesdames, messieurs les sénateurs, votre engagement pour introduire plus d'équité dans notre système de retraite.

Dès 2018, le Sénat s'est mobilisé pour travailler sur une réforme globale du système de retraite, avec plusieurs colloques et travaux auxquels j'ai eu le plaisir d'assister. Je cite la présentation

Ces trois objectifs sont au coeur des recommandations du Sénat sur les retraites depuis plus de vingt ans. » Je ne puis qu'être d'accord avec ces trois objectifs. Et je veux saluer les travaux, toujours d'une grande qualité, produits par votre assemblée je pense notamment aux rapports de M. René-Paul Savary, dont chacun connaît ici l'investissement et la maîtrise du sujet. Les petites pensions de retraite sont une préoccupation du Gouvernement. Je veux rappeler que la réforme adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, avant la crise sanitaire, prévoyait ces mesures de justice sociale. Je veux aussi rappeler que j'avais pris l'engagement d'aller plus loin sur ce sujet. C'est pour cela que le Premier ministre a demandé aux députés Turquois et Causse de produire un rapport et des propositions. Ces travaux sont en cours. Ils nous permettront, j'en suis sûr, d'avoir une meilleure vision d'ensemble : conjoints collaborateurs, aides familiaux, mais aussi artisans et indépendants, salariés précaires, autant de nos concitoyens qui, eux aussi, perçoivent généralement des petites retraites après un parcours professionnel souvent difficile. Le texte qui vous est soumis n'est pas exhaustif, et soyez convaincus que le Gouvernement a bien l'ensemble du sujet en tête. Mesdames, messieurs les sénateurs, l'examen à l'Assemblée nationale a permis d'aboutir à un texte équilibré. L'article 1 porte sur la revalorisation des pensions agricoles. Il s'agit du coeur de cette proposition de loi. Il reprend la garantie d'une pension totale équivalente à au moins 85 % du SMIC net agricole pour les chefs d'exploitation ayant effectué une carrière complète.

2022. Je sais que certains souhaiteraient que cette mesure s'applique encore plus vite, et c'est compréhensible. Je veux donc rappeler quelques éléments, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale. Notre devoir, c'est de ne pas trahir la confiance du citoyen. En 2014, il a fallu seize mois pour la mise en place de la garantie à 75 % du SMIC. % du SMIC. Et vous savez bien, mesdames, messieurs les sénateurs, que cette garantie figurait déjà dans la loi Peiro, en 2002. Plus d'une décennie d'attente Aussi, je me refuse à faire voter des textes inapplicables, fussent-ils adoptés à l'unanimité. Voilà pourquoi le texte prévoit une application « au plus tard au 1 janvier 2022 Ne trahissons pas les attentes des agriculteurs et des agricultrices avec de fausses promesses. Cette proposition de loi est un texte de progrès. Plus de 200 000 personnes, en métropole et dans les outre-mer, bénéficieront d'une hausse moyenne d'environ 110 euros de leur pension de retraite chaque mois. J'ai parlé de l'outre-mer ; c'est le coeur de l'article 3. Le Gouvernement est conscient de la spécificité de l'activité économique sur ces territoires. C'est pourquoi le texte propose une adaptation de l'article 1 aux spécificités de carrière des agriculteurs ultramarins. Son application sera plus souple sur la durée d'affiliation et sur la durée cotisée, ce qui constituera un progrès. Ainsi, tous les retraités agriculteurs ultramarins qui ont liquidé à taux plein bénéficieront de la garantie. L'article 4 s'inscrit dans cette logique de progrès pour les territoires ultramarins, en élargissant la couverture des salariés agricoles en matière de retraite complémentaire. Enfin, s'agissant du financement, je veux rappeler aux parlementaires que ces débats auront lieu dans le cadre des lois budgétaires et à la lumière des travaux de la mission Causse-Turquois, que j'évoquais. Cette Cette proposition de loi nous le rappelle, beaucoup reste à faire pour offrir à tous nos concitoyens un système de retraite juste, pérenne et équitable. Je voudrais terminer par un rappel, car ce texte s'inscrit dans une histoire, celle d'initiatives parlementaires visant à garantir un meilleur niveau de vie aux pensionnés agricoles. Je pense à la proposition de loi qui permit la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. C'était au tournant du siècle dernier. Si bien des choses ont évolué depuis lors, les débats tournaient déjà autour de deux sujets : la faiblesse des pensions de nos agriculteurs au regard de leurs efforts et de leur place dans la société ; les difficultés de financement inhérentes à ce régime. Cette proposition de loi était issue du travail mené par le député Germinal Peiro. L'apport du Sénat, notamment à travers son rapporteur, le sénateur du Puy-de-Dôme Jean-Marc Juilhard, fut toutefois décisif. C'est lui qui porta l'inscription d'une garantie de pension fixée à 75 % du SMIC. Cette proposition de loi fut adoptée à l'unanimité et de façon conforme entre les deux chambres. En 2017, c'est un autre parlementaire du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, qui mit de nouveau ce sujet à l'agenda. Aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons l'occasion, tous ensemble, de permettre à des centaines de milliers de Françaises et de Français d'améliorer leur quotidien.

En 2016, quand nos collègues députés André Chassaigne et Huguette Bello ont déposé leur proposition de loi, ils prévoyaient son entrée en vigueur au 1 janvier 2018. Le texte que nous nous apprêtons à adopter devrait s'appliquer au 1 janvier 2022. Que de temps perdu pour arriver à cette mesure de justice, qui permettra de porter à 85 % du SMIC le montant garanti de pension pour un chef d'exploitation à carrière complète ! À l'heure où chacun s'attribue les mérites et la parenté de ce texte, nous n'oublions pas que le Gouvernement, ici au Sénat, avait fait échec à l'adoption définitive en première lecture de cette proposition de loi en 2018, en recourant au « vote bloqué Deux ans après, le Sénat reprend donc l'examen de ce texte qu'avait rapporté à l'époque notre ancien collègue Dominique Watrin. Je suis heureuse aujourd'hui de porter ce texte devant vous avec mon collègue René-Paul Savary. Je l'ai dit devant notre commission des affaires sociales et je le répète ici : ce texte est nécessaire, mais il n'est pas parfait, et, si nous allons le voter, nous n'oublions pas ses faiblesses. Je pense particulièrement à la question des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux, qui ne sont pas concernés par ce dispositif. Ce sont souvent des femmes avec de faibles pensions : il faudra que nous travaillions sur ce sujet, car c'est aussi un combat d'égalité, une question de justice et de reconnaissance du travail effectué. Je pense également au mécanisme d'écrêtement ajouté à l'Assemblée nationale, sur lequel nous avons une appréciation divergente avec mon collègue rapporteur. Je regrette qu'un tel dispositif vienne affaiblir cette avancée. Ces manques ne doivent cependant pas nous empêcher de voter ce texte et d'assurer au plus vite ce progrès social pour les exploitants agricoles retraités, actuels et futurs. Je vous parle d'avancées et je tiens à en souligner d'autres, que ce texte permet également. Nous sommes au Sénat et, vous le savez, nous nous devons de veiller à la bonne application de la loi sur l'ensemble de nos territoires. de nos territoires. Or, dans les départements d'outre-mer, la « garantie 75 % » n'était pas encore une réalité. Alors que les critères d'éligibilité prévus ne correspondent pas aux réalités des exploitations agricoles ultramarines, ce texte vient apporter des adaptations nécessaires, en aménageant notamment la prise en compte de la durée d'assurance. La « garantie 85 % » que nous allons adopter trouvera donc à s'appliquer dans l'ensemble des départements. Nous nous apprêtons également à renforcer les droits à la retraite complémentaire pour les salariés agricoles de la Guadeloupe et de La Réunion, pour qui elle n'existe pas encore. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte est important. Aussi, au nom de la commission des affaires sociales, nous vous invitons à le voter et à contribuer ainsi à compenser, pour les exploitants agricoles retraités, l'impact sur leurs pensions des faibles revenus qu'ils connaissent trop souvent durant leur carrière. Bravo ! La parole

et d'entreprise agricole qui ont fait leur carrière à temps complet, nous ne devons pas oublier que ce sont aussi les revenus des agriculteurs qu'il faut travailler à améliorer. Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, dans un système à points, de faibles revenus débouchent

le 21 décembre 2016, quelques mois avant l'élection présidentielle, donc dans un contexte budgétaire bien particulier, Huguette Bello et André Chassaigne déposaient à l'Assemblée nationale la proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui. Cosignée par les membres du groupe GDR, elle avait pour ambition de revaloriser les petites pensions de retraite des agriculteurs et de pointer la situation des retraités Cette proposition de loi s'articule autour de deux piliers. D'un côté, les articles 1 et 2 garantissent un niveau minimum de pension à l'ensemble des retraités, par une augmentation de leur montant à 85 % du niveau minimum du SMIC

les articles 3 à 5 contiennent des dispositions en faveur de la revalorisation des pensions des retraites agricoles dans les départements et régions d'outre-mer, en facilitant l'accès des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ultramarins à la garantie « 75 % du SMIC en garantissant la couverture des salariés agricoles par les régimes d'assurance vieillesse complémentaire sur l'ensemble du territoire national. La commission des affaires sociales du Sénat a adopté le 24 juin dernier, à l'unanimité et sans modification, cette proposition de loi de revalorisation des petites retraites agricoles. C'est bien là l'essentiel. Et cela démontre que, quel que soit notre bord politique, quel que soit notre territoire, quelle que soit l'époque, notre assemblée a toujours tenu en grande estime le monde agricole. Nous savons tous ce que la France leur doit et quel pilier ils constituent dans notre république. D'aucuns voudront nous rappeler le chemin chaotique de cette proposition de loi et transformer cette belle conclusion avec un regard politique qui me semble malvenu aujourd'hui, voire essayer de nous reprocher de voter aujourd'hui ce que nous aurions fait échouer hier À chacun sa vérité », aurait dit Luigi Pirandello. Mais il est essentiel malgré tout de rappeler ici quelques éléments factuels, qui permettront à chacun de bien comprendre nos décisions. Le texte, porté par le chef de file des élus communistes André Chassaigne, avait été adopté à l'unanimité en première lecture en février 2017, sous la précédente législature. En mai 2018, une procédure de vote bloqué, le Gouvernement a demandé au Sénat un report de la date d'application de cette proposition. Le groupe CRCE a préféré retirer ce texte plutôt que de voter cette modification.

Nous sortions des états généraux de l'alimentation, qui s'étaient clôturés seulement deux mois avant et avaient pour principal objectif de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Nous étions en pleine préparation d'une réforme systémique des retraites, dont l'ambition, en particulier pour le monde agricole, allait bien au-delà de la proposition que nous examinons aujourd'hui. Et avec quel succès ! Nous étions convaincus que cette proposition de loi, à l'époque, ne répondait pas à la nécessité d'agir avec réalisme, équité et l'assurance d'un financement pérenne.

choisie ! Vous êtes gonflé ! Au regard de cette réalité de l'époque, nous avions donc l'impression d'une loi construite dans l'urgence, qui entrait en collision avec les travaux du Gouvernement et qui risquait d'apporter plus de confusion que de solutions. ! Je vous rappelle également, mes chers collègues, que la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs étaient alors opposés à cette proposition de loi non financée, non pérenne et bien moins ambitieuse pour eux que les engagements vers lesquels nous allions dans la réforme systémique de notre système de retraite. La crise de la covid-19 vient de frapper de plein fouet notre pays. Une crise économique sans précédent s'abat sur nous. Même si nombre de décisions pour en limiter l'ampleur ont été prises avec justesse par le Gouvernement, le pragmatisme doit aujourd'hui l'emporter sur toute considération, que celle-ci soit idéologique ou centrée sur la certitude d'avoir raison. Il était donc de bon sens de suspendre notre réforme systémique des retraites. Comme il est d'évidence de dire et rappeler que l'urgence pour les agriculteurs est toujours la même. C'est pourquoi nous nous réjouissons que cette proposition de loi revienne en discussion dans notre assemblée. Nous saluons l'accord qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous sommes conscients, et devons le rappeler, que cette avancée constitue un petit pas, qui ne résout pas tout, en particulier la situation des conjoints des chefs d'exploitation ou des employés agricoles.

depuis la Seconde Guerre mondiale, nos agriculteurs ont contribué à construire notre autonomie et notre souveraineté alimentaire. Je veux à ce titre saluer leur mobilisation sans faille durant la crise que nous traversons. Sans eux, la continuité de la chaîne alimentaire n'aurait pas été garantie. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture était très attendue, tant en métropole que dans les territoires ultramarins. Elle vise à revaloriser

Cette mesure correspond à une demande formulée depuis 2003 par la profession agricole. Le Gouvernement a néanmoins souhaité reporter l'entrée en vigueur de cette disposition à janvier 2022, tout en restreignant le nombre des bénéficiaires potentiels- ils

Pour des raisons de justice sociale, il me semble que nous devons procéder à la revalorisation des retraites agricoles, et cela le plus tôt possible. En effet, le montant moyen des retraites s'élève actuellement à 905 euros- 953 euros pour les hommes et 852 euros pour les femmes. Le texte que nous examinons aujourd'hui le porterait à 1 025 euros. Depuis Depuis près de cinquante ans, le monde agricole a contribué à l'essor économique de notre pays. Force est de constater qu'il n'en a pas toujours tiré les bénéfices. Ce métier est beau, mais difficile. La fatigue est plus que réelle et les heures de travail ne se comptent pas. Est-il nécessaire de rappeler que l'élevage nécessite un investissement de 365 jours par an ?

Pour des raisons d'attractivité économique du métier et plus encore d'accès au foncier, de nombreux jeunes agriculteurs renoncent à s'installer. Il s'agit d'un véritable enjeu de transmission et de renouvellement des générations.

sujet sur lequel mon collègue Jean-Louis Lagourgue avait alerté le ministre de l'agriculture et de l'alimentation en février dernier. Cette mesure bénéficiera notamment aux retraités agricoles de Guadeloupe et de La Réunion, qui ne bénéficient pas d'accord leur facilitant cet accès, contrairement aux agriculteurs de Martinique et de Guyane. Nous saluons cette avancée importante, notamment pour les chefs d'exploitation. Très Très peu d'agriculteurs ultramarins arrivant à l'âge de la retraite peuvent faire état d'une carrière complète et bénéficier du dispositif de garantie de 75 % du SMIC. Les agriculteurs ultramarins retraités perçoivent en moyenne retraités perçoivent en moyenne 375 euros de pension et un quart d'entre eux perçoit moins de 100 euros. Aussi, nous accueillons très favorablement cette disposition. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera

nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer. Le report de la réforme des retraites nous offre l'occasion de reprendre là où nous en étions restés. Près de quatre ans après le dépôt de la proposition de loi ... Que de temps perdu pour le monde agricole ! La crise sanitaire que nous vivons éclaire d'un jour nouveau cette proposition de loi,

les agriculteurs ont démontré leur grand sens des responsabilités et leur capacité à s'adapter. Et toujours pour un revenu bien trop faible, ce qui est la source de tous leurs maux

Aussi, notre objectif collectif doit être de garantir une rémunération décente aux agriculteurs. Toutefois- faut-il le préciser ? -, le texte que nous examinons aujourd'hui n'est qu'une étape dans la revalorisation des professions agricoles. Son article 1 vise à augmenter le niveau de pension de base et complémentaire minimal des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, en le passant à 85 % du SMIC, soit un peu plus de 1 000 euros, ce qui le rapproche du seuil de pauvreté. Il s'agit d'une avancée importante, mais qui demeure à mon avis très incomplète. Elle est même quelque peu rabotée par rapport à son ambition initiale à la suite à son passage à l'Assemblée nationale il y a dix jours. En effet, les députés de la majorité ont adopté un mécanisme d'écrêtement en fonction du montant de retraite tous régimes confondus. Un retraité sur trois ne pourra donc pas bénéficier de la garantie minimale de retraite. L'argument avancé est de permettre l'équité entre les assurés monopensionnés et les assurés polypensionnés. En réalité, cela illustre une nouvelle fois que le travail agricole n'est pas reconnu à sa juste valeur.

Ces femmes ne sont pourtant pas moins méritantes que leurs conjoints. Elles sont même des maillons indispensables au sein des exploitations agricoles. Eh oui ! Sans remettre en cause l'avancée permise par cette proposition de loi, celle-ci risque de créer, dans le même temps, davantage d'inégalités. Aussi, j'invite le Gouvernement à combler cette lacune d'ici à la mise en oeuvre effective de cette loi. Pour cela, il faudra notamment amorcer la redéfinition du statut et des rémunérations des conjoints et des aidants familiaux. Enfin, je tiens à saluer les avancées permises par ce texte pour les agriculteurs des départements d'outre-mer qui subissent actuellement plusieurs inégalités. Pour une carrière complète, les non-salariés agricoles ultramarins perçoivent une pension moyenne d'environ 200 euros de moins qu'un retraité en métropole. Moins du quart des monopensionnés ultramarins du régime des non-salariés agricoles a réalisé une carrière complète. Par conséquent, rares sont les bénéficiaires de la garantie des 75 % du SMIC. Concernant le financement, le Gouvernement a levé le gage de la proposition de loi. L'article 2 qui instituait une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières a été supprimé afin de renvoyer la question du financement au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dont acte ! Nous serons au rendez-vous, à l'automne, pour finaliser ce dernier chapitre.

La situation des conjoints n'est toujours pas réglée ; il faudra s'y atteler urgemment. Malgré ces réserves, le groupe Union Centriste votera en faveur de cette proposition de loi pour enfin clore cette séquence engagée il y a près de quatre ans, c'est-à-dire le

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez rappelé l'histoire des retraites agricoles et des propositions de loi, auxquelles les gouvernements de l'époque ne s'étaient pas opposés, bien au contraire.

n'y a eu plus rien, si ce n'est la proposition de loi de notre collègue député André Chassaigne, que nous allions voter à l'unanimité, mais que le gouvernement auquel vous appartenez a bloqué de manière abrupte et même, disons-le, assez brutale.

Requier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les retraités agricoles d'aujourd'hui sont les agriculteurs d'hier, ceux qui ont accompagné la modernisation de notre agriculture après la guerre, ceux qui ont permis à la France de se hisser au rang de grande nation agricole dans un monde devenu de plus en plus compétitif. Les retraités agricoles de demain, ce sont les agriculteurs d'aujourd'hui, ceux qui s'engagent dans la transition écologique au service de l'intérêt général, ceux qui se sont investis sans relâche, en pleine crise sanitaire, pour garantir à nos concitoyens des étals fournis, incarnant ainsi une part de la souveraineté alimentaire que notre collègue du groupe du RDSE, Françoise Laborde, encourage fermement. nul besoin dans cet hémicycle de démontrer combien les agriculteurs contribuent à l'aménagement du territoire. Pour toutes ces raisons et en retour du rôle économique et stratégique incontournable du secteur agricole, toutes les femmes et tous les hommes qui l'animent méritent la garantie d'un revenu décent à la hauteur de leur engagement. Or le niveau de pension moyen des retraités agricoles est le plus faible de tous les régimes, malgré des ajustements au fil des années. Je pense par exemple à la loi dite du 4 mars 2002, qui, en instaurant le principe d'une pension à 75 % du SMIC par le biais de la retraite complémentaire obligatoire, a amélioré les droits des retraités agricoles sans toutefois parvenir à l'objectif chiffré. Je rappelle aussi le plan quinquennal de revalorisation mis en oeuvre en 2012 qui a mobilisé près de 900 millions d'euros. Plus près de nous, la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites a permis de faire bénéficier aux conjoints et aides familiaux des points gratuits de retraite complémentaire de manière rétroactive. Néanmoins, ces réformes n'ont pas permis de combler l'écart entre les différentes catégories de retraités. Le constat est unanime : voir nos anciens agriculteurs toucher, pour la majorité d'entre eux, une pension inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est plus tolérable. En 2017, le montant moyen de la pension de droit direct était de 700 euros il existait une inégalité criante entre les hommes et les femmes : 900 euros pour les premiers et 530 euros pour les secondes. Certes, nous connaissons les raisons structurelles de cette situation : des parcours de carrière discontinus, un effort contributif contributif pas toujours suffisant, un régime d'assurance vieillesse caractérisé par un fort déséquilibre démographique qui complique son financement. Plus globalement, comme l'ont souligné nos collègues rapporteurs, les faibles revenus produisent de faibles pensions. C'est pourquoi, en marge de ce débat, je souhaitais également souligner une autre nécessité sous-jacente au problème des retraites, celle de poursuivre le travail sur la question des revenus des exploitants. nous y sommes tous sensibles et nous devons continuer à encourager toutes les mesures allant dans le sens de prix véritablement rémunérateurs. En attendant, le groupe du RDSE soutiendra la proposition de loi de nos collègues députés. Je rappelle qu'il est depuis longtemps attentif aux retraités : ainsi, deux de ses membres ont déposé en 1998 une proposition de loi allant dans le sens d'une amélioration des pensions. nous appelons de nos voeux l'instauration d'une pension à 85 % du SMIC. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole se verront ainsi garantir un revenu mensuel de 1 000 euros. La proposition de loi porte également un intérêt à la situation des retraités ultramarins. Nous sommes sensibles à cette mesure d'équité dans des territoires qui ont des spécificités auxquelles il faut répondre afin de ne pas creuser l'écart entre l'hexagone et l'outre-mer. Parmi les regrets que nous sommes nombreux à partager, je tiens tout d'abord à évoquer les interrogations qui existent sur le sort des retraites en cours. Sans méconnaître les enjeux budgétaires, nous attendons des réponses sur ce que l'on appelle « le stock ». Ensuite, le texte laisse de côté la situation des conjoints collaborateurs ou aidants familiaux- je pense en particulier à la situation des agricultrices. Comme vous le savez, mes chers collègues, la délégation aux droits des femmes du Sénat s'est penchée en 2017

dont quelques-unes visaient à prendre en compte la situation des agricultrices retraitées qui sont placées plus souvent que les hommes dans des situations de précarité financière. Aussi, j'espère, monsieur le secrétaire d'État, que ce texte ne sera que le début d'une plus large réflexion sur l'avenir de tous les acteurs du monde agricole- salariés, conjoints et aidants. À ce stade,

Aussi, nous comptons sur vous, monsieur le secrétaire d'État, pour envisager des mesures dès 2021, plutôt qu'en 2022. Dois-je rappeler que la proposition de loi a été déposée en 2016 ? déposée en 2016 ? Le plus tôt sera donc le mieux ! Le monde agricole nous regarde. Nous avons tous suffisamment croisé de retraités en difficulté pour savoir qu'un effort de solidarité nationale à leur égard est une reconnaissance, une obligation et un devoir moral.

madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui répond à une nécessité et à une urgence sociale. Il est en effet indispensable de revaloriser les retraites des chefs d'exploitation agricole. Il existe des petites retraites dans d'autres professions, chacun le sait, mais c'est dans le secteur agricole qu'elles sont les plus faibles. Le montant moyen de la pension d'un retraité agricole se situe entre 700 euros et 800 euros en métropole et bien moins encore dans nos territoires ultramarins,

Cette situation contraint en effet nombre d'agriculteurs à poursuivre leur activité : 15 % de nos agriculteurs sont encore en activité, alors qu'ils ont plus de 65 ans- certains vont au-delà de 70 ans ... Cela contribue à retarder l'installation de jeunes, voire à les décourager un peu plus d'exercer ce beau, mais très difficile métier. Le principal problème des retraites agricoles réside dans la faiblesse des revenus professionnels. Sur ce point, malgré les très fortes attentes exprimées à l'occasion des états généraux de l'alimentation, la loi Égalim n'a malheureusement pas permis d'avancer. L'enjeu d'une meilleure répartition de la valeur entre les producteurs, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution reste devant nous, tout comme la nécessité d'une politique agricole commune qui protège les plus petits producteurs et garantit des revenus justes et stables aux agriculteurs. Néanmoins, sans attendre davantage- trop de temps a déjà été perdu ! -, chaque agriculteur doit pouvoir bénéficier d'une pension décente au moment où il cesse son activité. Il y va de la justice sociale comme de la promotion d'un certain type de modèle agricole. Si nous voulons une agriculture avec des agriculteurs- je rappelle que le porte-parole de la Commission européenne se demandait il y a quelques mois encore, si nous avions besoin d'autant d'agriculteurs en Europe si nous voulons résister aux phénomènes de financiarisation de l'agriculture et d'accaparement des terres agricoles, si nous voulons une agriculture à taille humaine, garante de qualité et de sécurité alimentaire, alors, il faut soutenir nos producteurs. est l'objet de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui qui vise à leur garantir un niveau minimum de pension supérieur au seuil de pauvreté. Ainsi, son article 1 porte le montant minimum des retraites agricoles à 85 % du SMIC net. Cette proposition de loi, loi, portée depuis 2016 avec détermination par notre collègue et ami, le député André Chassaigne, arrive au bout du circuit parlementaire après de nombreuses péripéties. Je rappelle que, en 2017, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté ce texte à l'unanimité, mais, par un artifice procédural, le Gouvernement en a finalement empêché l'adoption. Nous espérions que l'exécutif avait retrouvé le sens de l'intérêt général à la faveur de cette nouvelle occasion. C'était sans compter l'adoption d'un amendement, par La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui tend à réduire la portée de ce texte et à en retarder l'application. Je vous ai bien écouté, monsieur le secrétaire Vous essayez de vous rattraper, en évoquant janvier 2022 « au plus tard », mais je vous le dis clairement : le plus tôt sera le mieux ! La majorité présidentielle a modifié la proposition de loi initiale, en instaurant un dispositif d'écrêtement qui tourne le dos au principe d'universalité des retraites. En introduisant une distinction

Pis, cette mesure, défendue par la majorité présidentielle, va exclure 100 000 personnes du bénéfice du dispositif, soit le tiers des bénéficiaires potentiels. Le monde agricole mérite pourtant un geste fort de reconnaissance. Il a encore démontré durant la crise sanitaire son caractère stratégique, et les agriculteurs ont fait preuve d'un dévouement que les Français, eux, ont reconnu. Cela dit, Cela dit, ce texte est une première étape vers la revalorisation des pensions de retraite du monde agricole. Il nous faudra poursuivre le travail en faveur des conjoints collaborateurs, c'est-à-dire généralement des femmes, ou encore des aides familiaux, car leurs pensions, loin de refléter leur rôle

Nous mettions tous unanimement en exergue la nécessité d'une meilleure retraite pour nos agriculteurs. Tous, sauf le Gouvernement qui a préféré nous mettre au pied du mur avec la technique parlementaire du vote bloqué pour ne pas permettre la revalorisation immédiate et nécessaire que nous souhaitions. Nous voilà enfin de retour aujourd'hui pour reprendre la discussion sur ce texte essentiel pour le niveau de vie de nos retraités, qui n'ont pas aujourd'hui le juste retour du labeur de toute une vie. Georges Pompidou, Président de la République, qui connaissait bien la ruralité du Cantal et la rudesse de la vie des agriculteurs, ainsi : « Mon père et ma mère appartenaient profondément à la famille française, dure au travail, économe, croyant au mérite, aux vertus de l'esprit, aux qualités du coeur. Je n'ai pas eu une enfance gâtée, mais si loin que je remonte je n'ai reçu que des leçons de droiture, d'honnêteté et de travail. Il en reste toujours quelque chose Ce propos résonne toujours fortement pour nous, fils et petit-fils de paysans, car nous sommes plusieurs dans ce cas au sein de la Haute Assemblée. Nous avons tous été marqués par la retraite de misère de nos parents et grands-parents, et nous ne pouvons plus accepter le sort de nos nombreux retraités agricoles. J'en appelle à la dignité pour nos agriculteurs. J'en appelle à plus de justice pour nos territoires ruraux. J'en appelle à l'équité et à la solidarité des parlementaires pour des hommes et des femmes qui ont travaillé durement toute leur vie et qui se retrouvent, pour certains d'entre eux, sous le seuil de pauvreté Après le vote bloqué imposé par le Gouvernement, j'avais, avec mon éminent collègue Laurent Duplomb, déposé une proposition de loi similaire, car nous ne pouvions pas nous résigner. La dignité d'une nation se mesure aussi à l'aune de la considération qu'elle porte à ses aînés. La ténacité et le pouvoir de persuasion au plus haut niveau du « compagnon Dédé » font que cette proposition de loi est de nouveau discutée dans un contexte où la réforme globale des retraites est suspendue. Je ne puis que saluer ce retour.

sociales diverses ni la solidarité nationale, alors que les enfants accompagnent bien souvent leurs parents et leurs grands-parents en fin de vie à domicile. Cette préoccupation a été celle de gouvernements successifs depuis 2002.

85 %, c'est un minimum vital ! Il est essentiel que cette revalorisation à 85 % s'applique pour tous les retraités dès à présent. Le texte prévoit une revalorisation pour les actifs au 1 janvier 2021, et pour tous les retraités actuels en 2022. La nécessité d'une application immédiate pour tous, exprimée voilà deux ans, est toujours la même. Nos retraités ne peuvent pas attendre 2022 ! L'urgence était déjà présente hier, elle s'est même renforcée avec la crise financière de la covid, durant laquelle nos agriculteurs ont répondu présents en assurant notre approvisionnement et notre indépendance alimentaires

sociale agricole, la MSA, a précisé la semaine dernière que la chose était possible dès janvier 2021. Alors, allons-y ! Par ailleurs, les épouses et conjointes collaboratrices des agriculteurs doivent être incluses dans la réforme. Il serait totalement injuste que leur investissement au côté de leur conjoint ne soit pas pris en compte et considéré.

Je ne peux pas, avoir, d'un côté, des agriculteurs qui n'ont pas de retraite, et, de l'autre, un statut de cheminot et ne pas le changer. » Nous sommes aujourd'hui en 2020 et nous discutons pour la seconde fois de ce texte. Vous ne m'entendrez pas dire qu'une revalorisation peut se faire d'un claquement de doigts. Avouez, néanmoins, que vous n'avez rien fait pour accélérer cette dernière, et ce n'est rien de le dire. Il y a tout d'abord eu votre amendement reportant à 2020 cette revalorisation, alors que nous souhaitions, ici même au Sénat, qu'elle entre en vigueur dès 2019. Puis, il y a eu un vote bloqué pour nous en empêcher.

à préciser que nous parlons bien d'une revalorisation de pensions de retraite de 75 % à 85 % du SMIC. Il me faut souligner, et même marteler, que, aujourd'hui, un agriculteur sur trois à une retraite inférieure à 350 euros par mois. S'il y a bien une leçon que nous devons tirer du confinement, c'est que notre indépendance alimentaire est ô combien précieuse. Ces femmes et ces hommes répondent à nos besoins primaires. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont pris conscience que rien n'apparaît par magie dans les rayons des supermarchés. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer la retraite indécente de nos agriculteurs. Personne ne peut, non plus, ignorer la dureté de ce travail. Rendez-vous compte : alors que notre pays compte plus de 3 millions de personnes sans emploi, les maraîchers des Bouches-du-Rhône ont dû faire appel à des travailleurs détachés, car il n'y avait pas suffisamment de main-d'oeuvre. Comme souvent, je regrette la méthode du Gouvernement, pour des considérations non pas procédurales, mais plutôt politiques. Quand vous vous félicitez, dans les médias, de cette revalorisation, je ne suis pas sûre que vous mesuriez bien l'espérance que vous faites naître. Je regrette de ne pas avoir beaucoup entendu votre collègue Marlène Schiappa concernant la retraite des conjoints. En effet, les conjoints sont très souvent des conjointes, et leurs pensions resteront, quant à elles, à 550 euros par mois.

En effet, cette revalorisation ne concerne que les chefs d'exploitation. Cette autosatisfaction est indécente. Après autant de mobilisation, daigner porter à 85 % du SMIC la retraite d'une partie seulement

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, la commission n'a pas la même lecture que le Gouvernement de cet article, et particulièrement de son II. Nous l'avons constaté lors de l'audition de M. le secrétaire d'État pour préparer cette deuxième lecture. L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour que l'application du I se fasse au plus tard au 1 janvier 2022, et non plus nécessairement

Ainsi, soyons clairs, que vous le vouliez ou non, ce que dit le texte de loi dont nous débattons, c'est bien que vous pouvez avancer l'entrée en vigueur du II, et non du I, de l'article 1. Cela signifie que, dans le cas où le Gouvernement prendrait un décret anticipant la date du 1 janvier 2022, cette disposition n'aurait de valeur que pour les nouveaux retraités de l'Hexagone. Pour les retraités actuels, comme pour les adaptations retenues pour les agriculteurs des départements d'outre-mer, la date d'entrée en vigueur est précisée clairement dans la loi : ce sera le 1 janvier 2022 ! L'absence de coordination ne vous laisse donc pas la possibilité d'anticiper. Vous nous avez indiqué que si, d'aventure, vous décidiez d'anticiper l'entrée en vigueur, vous prendriez une circulaire permettant d'intégrer les retraités actuels et les outre-mer. C'est là une bien singulière interprétation de la hiérarchie des normes, que nous ne pouvons pas nous permettre de partager dans cette assemblée. Monsieur le secrétaire d'État, nous n'avons pas amendé ce texte pour ne pas retarder son adoption définitive. Aussi, notre souhait est de voir ces coordinations assurées dans un texte prochain, peut-être celui qui assurera le financement de cette réforme.

d'une allocation différentielle qui porte sur les retraites obligatoires, mais complémentaires, et qui ne sont pas dans le champ du PLFSS aujourd'hui. Vous aviez proposé de le faire dans

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, comme beaucoup ici, je viens d'un département où des hommes et des femmes ont participé fortement, et souvent durement, à relever la France, à une époque où l'on croyait encore à l'agriculture pour assurer notre indépendance alimentaire.

! Depuis lors, le mouvement de disparition des petites exploitations familiales s'est poursuivi. Il faut savoir que près de 100 000 emplois d'exploitants et d'ouvriers agricoles ont été perdus dans ma région

l'ont dit, un tiers des agriculteurs perçoivent moins de 350 euros par mois. Dès lors, ce dispositif de revalorisation des retraites à 85 % du SMIC, soit un peu plus de 1 000 euros, constitue une avancée juste et nécessaire pour celles et ceux qui ont tant donné pour relever notre agriculture. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de cette mesure avant 2022 est très importante, monsieur le secrétaire d'État. Dès lors, quand la majorité repousse l'application d'un an, au 1 janvier 2022, en faisant valoir des « motifs techniques », cela s'apparente à une triste et piètre diversion, d'autant que le président national de la MSA, M. Cormery, a bien indiqué qu'il n'y avait aucun obstacle de ce type qui empêchait une entrée en vigueur du dispositif dès le 1 janvier prochain. Je rejoins donc les positions de nos rapporteurs, et j'ose espérer que le Gouvernement

largement attendu dans les campagnes et par les plus fragiles de ceux qui tentent de vivre de la terre. Derrière la question des faibles retraites, par définition,

ensuite la démonstration d'une certaine mesquinerie, passez-moi le terme, à ne pas vouloir rendre justice immédiatement pour faire quelques économies. J'attire votre attention, mes chers collègues,

question. Vous décidez de faire l'économie d'une année, comme ma collègue Monique Lubin l'a fort bien dit, parce que vous avez besoin de temps. En revanche, pour supprimer l'ISF, vous n'avez pas eu besoin de temps, puisque vous l'avez fait quasi immédiatement !

dit qu'il peut, si vous prenez le bon décret, agir rapidement. Autre point sensible, vous visez les plus faibles. En disant que les polypensionnés vont être écrêtés, on a l'impression que l'on va agir sur des riches parmi les retraités agricoles. Pensez donc, des polypensionnés ... Mais pourquoi le sont-ils ? Parce qu'ils n'ont pas assez de revenus sur leur exploitation et qu'ils sont obligés d'aller chercher des revenus à l'extérieur pour compléter

quelle était votre philosophie dans cette histoire d'écrêtement. Le Gouvernement considère qu'il s'agira d'une allocation complémentaire, en quelque sorte de solidarité, et que, comme toute allocation de solidarité, elle doit tenir compte de tous les revenus. Il faut donc qu'il y ait une somme maximale à ne pas dépasser. Toutefois, ne pourrait-on pas considérer, puisque l'on parle là d'agriculteurs qui auront travaillé et cotisé une carrière pleine,

donc ne pas appliquer d'écrêtement ? Je le répète, dans aucune autre profession nous ne pratiquons les écrêtements de pension de retraite. Je demande réellement à ce que l'on y réfléchisse, non pas cette fois-ci, nous l'avons bien compris, mais dans des temps très proches.

Le minimum que l'on puisse faire est de voter ce texte et de penser, surtout, à son financement, qui ne devrait pas tarder. On va encore parler de la dette sociale dans quelques jours. Tout cela est lié et nous renvoie à des ruptures d'égalité tellement flagrantes, monsieur le secrétaire d'État, que je me demande combien de temps encore nos concitoyens pourront les supporter.

afin que cette revalorisation puisse se faire sans délai. Par un artifice de procédure, à savoir un vote bloqué, que peu d'entre nous connaissaient, nous n'avons pas pu le faire. Nous avons été empêchés, tous ici, pour des raisons purement politiciennes, parce que, aujourd'hui, c'est votre texte que vous présentez. C'est à votre bénéfice, effectivement, que vous souhaitez que cette loi puisse passer. Que de temps perdu ! Je suis élue d'un département agricole. En Gironde,

je ne reviendrai pas sur les vicissitudes qu'a connues ce texte, mais je voudrais insister sur quelques points. Tout d'abord, je tiens à dire que les retraités agricoles sont étroitement liés aux actifs agricoles. Pour qu'il y ait des actifs agricoles, il faut que celui qui cesse son activité sacrifie une partie de ses biens, de son patrimoine, afin que son successeur puisse y arriver. Vous savez tous quelles sont les difficultés

Les retraités agricoles, souvent, lorsqu'ils ont la chance d'avoir des enfants qui leur succèdent, se sacrifient encore un peu, comme vient de le dire ma collègue. Il est très important d'avoir cette réalité donc la moindre des choses que de leur donner ces quelques euros que nous sommes en train de voter. Nous ne sommes pas en train de voter quelque chose d'exceptionnel ; nous sommes simplement en train d'offrir une retraite de 1 000 euros à des gens qui ont travaillé toute leur carrière.

elles n'ont pas toujours beaucoup cotisé. Certes, il y a eu quelques problèmes de cotisation, mais la tâche a été accomplie. Le revenu était celui du ménage et il était faible. C'est aussi pour cette raison que les cotisations n'ont pas été payées

et syndicaux. La portée de ce texte a été réduite par la majorité présidentielle de l'Assemblée nationale ; cela laisse tout de même un goût amer chez les retraités, tant leurs pensions restent faibles : certains d'entre eux ne cotisent même pas suffisamment

et sa capacité à se montrer constant dans ses travaux. Nous continuerons donc à défendre la nécessité d'une revalorisation de toutes les pensions de retraite agricoles, en particulier celles des femmes.

prévu de donner : « Dans ce que l'on appelle les outre-mer, un chef d'exploitation agricole monopensionné sur deux perçoit une retraite inférieure à 333 euros par mois. Cela s'explique par notre histoire particulière, notamment l'arrivée tardive des caisses de retraite agricole dans nos territoires. « Le texte que nous nous apprêtons à voter leur offre la garantie d'une pension à 85 % du SMIC. Cela représente une avancée considérable pour eux à partir de 2022- enfin ! -, ils passeront au-dessus du seuil de pauvreté. « Je regrette le temps perdu depuis la première lecture de ce texte, ainsi que l'exclusion des polypensionnés du bénéfice de cette mesure, mais je salue la suppression, pour les agriculteurs desdits outre-mer, de la condition d'affiliation de 70 trimestres. « Cette décision vient quelque peu réparer l'histoire ; je tiens, même si je ne peux être présente, à avoir une pensée pour tous ces travailleurs besogneux qui ont trop longtemps vécu dans la misère.